Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Travail et emploi

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le budget de la mission « Travail et emploi » pour 2018, premier du quinquennat, est un budget de transformation.

Oui, le Gouvernement souhaite manifestement rompre avec la logique inflationniste poursuivie sous le quinquennat précédent, dont les résultats sont pour le moins mitigés. La mesure la plus commentée est certainement la réduction de l'enveloppe des emplois aidés. Seuls 200 000 contrats dans le secteur non marchand seront, en effet, conclus en 2018. Bien évidemment, je ne conteste pas l'utilité de ces emplois pour les collectivités territoriales et pour les associations. des études et des statistiques, la DARES, le taux de retour à l'emploi des bénéficiaires d'un contrat aidé dans le secteur non marchand n'est que de 41 %. Pis, les contrats aidés seraient à l'origine d'un « effet stigmate », diminuant l'employabilité de leurs bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle, lors de l'examen des projets de loi de finances pour 2015 et 2016, le Sénat a proposé de diminuer le nombre d'emplois aidés, considérant, à raison, que ceux-ci constituaient une réponse de court terme, souvent motivée par des raisons purement statistiques, au problème du chômage. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de ne pas reconduire certains dispositifs, tels que l'aide à l'embauche à destination des PME, créée en 2016 et opportunément prolongée jusqu'en 2017 par le précédent gouvernement. La pérennisation de cette aide aurait conduit à un important effet d'aubaine, alors que son coût pour les finances publiques était compris entre 3 et 4 milliards d'euros. Des efforts seront, en outre, demandés aux opérateurs, notamment Pôle emploi, qui verra le montant de sa subvention diminuer de 50 millions d'euros. Enfin, le ministère du travail prendra toute sa part de l'effort de réduction des déficits, comme il l'a fait au cours des années précédentes.

ce budget est l'efficacité. C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures, dit-on. Force est de constater que cela n'est pas le cas en matière de politique de l'emploi ! C'est pourquoi, à des mesures de court terme, le Gouvernement a préféré un plan ambitieux d'investissement dans les compétences, qui comportera deux volets d'une part, la poursuite de la montée en puissance de la garantie jeunes- 160 millions d'euros seront ainsi versés aux missions locales pour assurer l'accompagnement de 100 000 jeunes ; d'autre part, la mise en place d'un plan de formation à destination des demandeurs d'emploi faiblement qualifiés et des jeunes décrocheurs. Au total, 2 millions d'actions de formation devraient être proposées sur le quinquennat. Le Gouvernement a également souhaité s'attaquer à la question du chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en relançant l'expérimentation des emplois francs, selon des modalités différentes de celles qui avaient été retenues en 2013. La situation économique et sociale de ces quartiers me semble justifier un tel dispositif, auquel je souhaite que nous donnions une chance. Le troisième axe de ce budget est la sincérité. La décision prise à l'été 2017 de redimensionner l'enveloppe de contrats aidés n'était pas facile à prendre. Certains l'ont qualifiée, à juste titre, de « brutale », mais il s'agissait de répondre dans l'urgence à un risque de dérapage budgétaire identifié par la Cour des comptes dans son audit des finances publiques. Je rappelle, à cet égard,

D'aucuns ont dénoncé l'irresponsabilité du Gouvernement. Toutefois, l'irresponsabilité n'était-elle pas du côté du précédent gouvernement, qui a poussé les collectivités à recruter massivement, conduisant à ce que 70 % de l'enveloppe votée en loi de finances initiale soit consommée dès le premier semestre 2017 ? L'irresponsabilité aurait été de laisser faire, en bafouant le vote du Parlement. Comme chaque année, notre assemblée aurait dénoncé le dérapage inacceptable lié au dépassement de l'enveloppe de contrats aidés. Je rappelle, pour mémoire, que, en 2016, la dépense en faveur des contrats aidés avait été supérieure de plus de 1 milliard d'euros aux prévisions. Pour 2018, les choses sont claires et le choix du Gouvernement de se tenir à l'enveloppe votée par le Parlement permettra d'améliorer la sincérité du budget. J'espère, d'ailleurs, madame la ministre, que le Gouvernement se tiendra à cette enveloppe, ce qui n'a vraiment pas été le cas par le passé. Mes chers collègues, le budget qui nous est proposé se concentre donc sur l'essentiel : améliorer l'employabilité des personnes les plus éloignées du marché du travail. Des choix clairs de politique publique y sont exprimés, au prix, il est vrai, de la non-reconduction de dispositifs dont l'efficacité statistique est indéniable, mais dont l'impact sur le marché du travail est faible. Aussi, mes chers collègues, la commission des finances s'est-elle prononcée en faveur de l'adoption des crédits de la mission « Travail et emploi » et du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame, chers collègues, la mission « Travail et emploi » regroupe les moyens consacrés à la politique de l'emploi. L'évolution de ses crédits a donc des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de Français. force est de constater que cette mission est, avec celle qui réunit les crédits du logement, l'une des deux sacrifiées du projet de loi de finances pour 2018. Ce budget va fragiliser nombre de demandeurs d'emploi et de personnes précaires, alors que le taux de chômage demeure très élevé- il atteignait 9,5 % au deuxième trimestre 2017 -et qu'il est surtout très inquiétant pour les publics les plus éloignés de l'emploi, il n'a cessé de croître. Je pense notamment au taux d'emploi des seniors, qui demeure faible. À périmètre constant, la diminution des crédits de la mission sera record : elle atteindra plus de 4 milliards d'euros en autorisations d'engagement et plus de 2 milliards d'euros en crédits de paiement. Ce budget est donc un mauvais coup pour les personnes les plus fragiles. La diminution du nombre de contrats aidés en est probablement l'exemple le plus emblématique. Pourtant, la décision brutale prise à l'été 2017 de réduire l'enveloppe de ces contrats, qui s'est traduite par d'importantes difficultés pour les collectivités territoriales et les associations, mais aussi dans de nombreuses écoles, à quelques semaines de la rentrée scolaire, a bien montré l'utilité de ces derniers, sans parler de la détresse dans laquelle des bénéficiaires non reconduits ont été jetés. Ces contrats constituent des instruments importants pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. En leur absence, la plupart des personnes concernées n'auraient tout simplement pas eu accès au marché du travail. La baisse prévue dans le présent budget a donc déjà conduit et conduira encore à une fragilisation de certains services publics. Elle aura des conséquences sociales importantes. En outre, le taux moyen de prise en charge par l'État étant revu à la baisse, passant de 72,1 % à 50 % du SMIC brut de 72,1 % à 50 % du SMIC brut entre 2017 et 2018, certaines structures associatives auront plus de difficultés à s'engager dans le dispositif des contrats aidés. De plus, cette baisse drastique jette l'opprobre sur les collectivités territoriales, qui ont été soupçonnées de tirer profit de l'effet d'aubaine provoqué par ce dispositif

Par ailleurs, le présent budget porte un coup aux actions en faveur de l'amélioration des conditions de travail, avec la baisse du montant de la subvention versée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, alors que l'Organisation mondiale de la santé estime que 1 euro dépensé dans le domaine de la santé au travail se traduit, pour les entreprises, par une économie de 13 euros. 13 euros. La poursuite de la réduction des effectifs de l'inspection du travail est elle aussi dommageable, surtout dans le contexte de la multiplication des sources de droit bientôt mise en place avec la mise en oeuvre des ordonnances le budget qui est soumis à notre examen est révélateur de l'incohérence de la politique menée par le Gouvernement, qui souhaite relancer l'apprentissage et, « en même temps », supprime l'aide financière en faveur des jeunes apprentis, qui lance un grand plan d'investissement dans les compétences et, « en même temps », diminue les crédits consacrés aux opérateurs chargés, sur le terrain, d'aider et d'accompagner les demandeurs d'emploi. Ainsi, la subvention pour charges de service public versée à Pôle emploi diminuera de 50 millions d'euros,

En outre, ce rapport précise que « les demandeurs d'emploi de longue durée sont sous-représentés dans l'accompagnement renforcé ». Que dire de la division par deux des crédits consacrés aux maisons de l'emploi ? Il semble que l'on crée les moyens de leur suppression par la diminution progressive de leur subvention. Le Gouvernement veut poursuivre la généralisation de la garantie jeunes et « en même temps », il ne réévalue pas sa contribution au financement des missions locales, alors que celles-ci devront accompagner près de 15 000 jeunes supplémentaires et que nombre de ces structures font face à une instabilité chronique de leurs financements, liée au retrait des financeurs locaux. Concernant le plan d'investissement dans les compétences, présenté par le Gouvernement comme l'alpha et l'oméga de sa politique de l'emploi, je constate que l'effort réel est bien inférieur au montant mis en avant dans la communication gouvernementale, tant sur le nombre de personnes formées que sur les moyens dégagés. En effet, dans la mesure où les crédits consacrés à la garantie jeunes et au « plan 500 000 formations » figuraient déjà dans le périmètre de la mission « Travail l'effort consenti ne s'élèvera qu'à 750 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 430 millions d'euros en crédits de paiement. En outre, des questions demeurent en suspens s'agissant du financement de ce plan et des moyens humains qui y seront consacrés.

Mes chers collègues, le budget 2018 de la mission « Travail et emploi » n'est pas un bon budget. Sa dynamique baissière sera aggravée au long des prochaines années par le projet de loi de programmation des finances publiques, qui prévoit une diminution de 17 % de ses crédits entre 2018 et 2020.

malgré une diminution de ses crédits de l'ordre de 1,5 milliard d'euros à périmètre constant, je partage la philosophie de la mission « Travail et emploi », qui consiste à mettre l'accent sur la formation continue plutôt que sur les dispositifs correctifs.

Pourtant, la qualification par les formations initiale et continue est, à mon sens, le meilleur vaccin contre le chômage de longue durée. Deuxième observation, les collectivités territoriales et les associations ont besoin de connaître, ne serait-ce qu'à grands traits, le volume des contrats aidés pour les années à venir, les secteurs prioritaires ainsi que le taux de prise en charge par l'État. Ce manque de visibilité fait régner un climat malsain, qui démobilise les acteurs publics et associatifs dans nos territoires. professionnelle des adultes doit bâtir rapidement un modèle de développement ambitieux et robuste pour retrouver un second souffle après des années de déclin. Malgré sa transformation en établissement public, l'AFPA est toujours dans un état critique. J'espère que son nouveau président saura fixer un nouveau cap stratégique. Le challenge, pour l'AFPA, est de créer une nouvelle dynamique, malgré une pyramide des âges défavorable et une culture interne qui n'a pas su s'adapter aux mutations de notre société. l'expérimentation des emplois francs, décidée dans la précipitation, pourrait entraîner un coût exorbitant pour les finances publiques, alors que son efficacité est douteuse et que ses modalités pratiques n'ont pas été communiquées au Parlement. Nous y reviendrons lors de la présentation de l'amendement de la commission Avant de conclure, je voudrais vous faire part, madame la ministre, de trois sujets d'inquiétude. Tout d'abord, la dette de l'UNEDIC atteint un niveau excessif : elle dépassera, à la fin de l'année 2018, 37 milliards d'euros, soit une année de ses recettes. Ce fardeau de la dette doit être combattu, car il risque, à terme, de pénaliser nos concitoyens les plus fragiles si les taux d'intérêt remontent brutalement. Il appartient au Gouvernement de mobiliser les partenaires sociaux Ensuite, toute proposition visant à un rapprochement, voire à une fusion entre les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat doit être examinée avec une extrême prudence, car l'on doit préserver les spécificités de l'artisanat. Enfin, la revalorisation du rôle des branches professionnelles ne doit pas aboutir à remettre en cause les prérogatives des régions en matière de pilotage de l'apprentissage. En conclusion, suivant mes recommandations, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission, sous réserve de l'adoption de son amendement sur les emplois francs, et un avis favorable à l'adoption du compte d'affectation spéciale relatif à l'apprentissage. Mes chers

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment pas, lors de la discussion de ce premier budget du quinquennat, évaluer l'action du Gouvernement ni lui faire un procès d'intention. On le sait, une politique du travail et de l'emploi se mesure essentiellement dans la durée. Notre groupe a soutenu les orientations de la politique de votre gouvernement, madame la ministre, en votant la loi d'habilitation des ordonnances. Nous attendons avec intérêt les lois sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Venons-en à votre budget. Il suscite, chez nous, quelques interrogations.

Je m'attarderai plus longuement sur les acteurs de la politique de l'emploi, les contrats aidés et les aides à l'emploi. Le constat du morcellement du service public de l'emploi est unanimement partagé. Il existe trop de structures, ce qui conduit à un manque de visibilité et à un inévitable gaspillage d'argent public. Je considère, pour ma part, qu'il est nécessaire de territorialiser beaucoup plus qu'aujourd'hui la politique de l'emploi, afin qu'elle soit au plus près des réalités du terrain. Les besoins ne sont pas les mêmes à Arras, à Marseille ou à Strasbourg. C'est pourquoi les structures qui en ont la charge doivent connaître la situation et les besoins de l'emploi dans leur périmètre et anticiper les mutations économiques. Elles doivent être actrices du développement local de l'emploi, en accompagnant les entreprises qui recherchent des salariés- parfois vainement. Ces missions sont celles des maisons de l'emploi. je connais bien ces structures, qui représentent, selon moi, l'outil le plus adapté pour orienter efficacement les politiques de l'emploi. La raison principale est qu'elles réussissent, là où elles existent, à mettre autour de la même table tous les acteurs

La raison avancée par Mme la ministre est la montée en puissance de Pôle emploi, ce qui peut s'entendre du point de vue du Gouvernement. Je dis, pour ma part, que les deux structures sont complémentaires. Pôle emploi se concentre sur les prestations de l'État en matière d'accès et de retour à l'emploi, quand les maisons de l'emploi doivent fédérer toutes les autres structures afin d'améliorer l'efficacité afin d'améliorer l'efficacité de leur gestion, ainsi que des dispositifs d'insertion et de lutte contre le chômage. Dans cet esprit, l'impératif serait plutôt de fusionner les plans locaux pour l'insertion et l'emploi et les missions locales- j'en préside une également -au sein des maisons de l'emploi. Par conséquent, je soutiendrai, avec nombre de mes collègues, les amendements visant à rétablir au niveau de 2017 les crédits des maisons de l'emploi. aborder l'épineuse question des contrats aidés. Vous décidez de financer, l'an prochain, 200 000 contrats aidés dans le secteur non marchand, tout en diminuant le taux de prise en charge par l'État. L'annonce de cette mesure a été mal reçue cet été, en raison, me semble-t-il, d'un défaut de pédagogie et d'un excès de précipitation. Il faut, en la matière, que l'on clarifie l'objectif

Les contrats aidés ne sont une bonne solution en matière d'accès à l'emploi que s'ils sont accompagnés d'une formation solide qualifiante. Sinon, il ne s'agit que d'emplois précaires sous perfusion d'argent public. Tout le monde partage

que le Gouvernement souhaite expérimenter, sur l'initiative d'une partie des députés de la majorité présidentielle. Il ne s'agit certes que d'une expérimentation, mais je partage les inquiétudes de notre rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales sur le coût de ce En la matière, je suis plutôt partisan de dispositifs comme la garantie jeunes, dont je salue la montée en puissance l'année prochaine. Plutôt qu'un emploi subventionné, il s'agit d'un parcours d'accompagnement vers l'emploi fondé sur des obligations et des engagements et des engagements réciproques entre le jeune bénéficiaire et la structure d'accompagnement qu'est la mission locale. Les contrats aidés ont été considérés par de nombreux élus et par les gouvernements précédents comme une aide aux collectivités publiques et aux associations. Une diminution a conduit à des réactions virulentes. Il est vrai que les collectivités territoriales ont de plus en plus de difficultés à assumer les missions qui leur sont transférées. C'est ce que traduit la Mais la solution doit être adaptée et ne peut reposer sur le dévoiement d'un dispositif conçu initialement pour lutter contre le chômage. C'est une question de cohérence. Il faudra,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est à la fois avec beaucoup de gravité et d'humilité que je prends part à ce débat sur la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances pour Ce débat place immédiatement le Gouvernement face à ses responsabilités et à ses engagements de campagne. Gravité ? Oui, la situation toujours plus préoccupante sur le front de l'emploi oblige à la gravité. Pourtant, si j'écoute Bruno Le Maire, nous sommes en passe d'être sauvés par une reprise ferme et solide. Si la reprise est là, elle me semble néanmoins fort timide et ne permet pas, en tout état de cause, d'améliorer durablement, à elle seule, la situation de l'emploi. Nous le savons, en dessous de 1,5 % de croissance, le rebond automatique et providentiel attendu en matière d'emploi n'a pas lieu. C'est donc à la structure du marché qu'il faut que nous nous attaquions. En cela, je trouve la philosophie du Gouvernement intéressante. Elle consiste à favoriser la prise d'initiatives, à libérer les énergies pour créer les emplois de demain et, « en même temps », à protéger les plus faibles dans des périodes dévastatrices sur le plan personnel.

un discours bien éloigné de la simplification outrancière, de la réduction de la pensée et de la politique-spectacle. Oui, il nous faut accompagner l'individu en tant qu'être humain, et non en tant que numéro, vers une formation sur ce point -, au plus près du terrain, au plus près des bassins d'emploi, au plus près des forces vives de nos territoires, donc des entreprises. Il nous faut être acteurs de cette grande mutation. Il nous faut remettre le travail au coeur de notre société. Si nous restons de simples spectateurs, alors la France demeurera un pays sous perfusion. Il nous faut avoir un temps d'avance sur les métiers et sur l'entreprise de demain, un temps d'avance sur l'accompagnement des jeunes et un temps d'avance dans la prise en charge des personnes en reconversion. Votre premier budget, madame la ministre, trace une perspective autour de laquelle sera articulé ce quinquennat. Si je salue votre façon de travailler avec les syndicats, qui nous fait entrer dans une forme de dialogue social qui répond aux enjeux du XXI siècle-

La politique de l'emploi ne peut pas se concevoir uniquement dans les ministères. Une connaissance aiguë du tissu économique est primordiale. Et qui sont les mieux placés, les plus compétents, les plus à même de travailler à la définition des emplois adéquats par bassin d'emploi que les acteurs locaux ? Il Il nous faut, à travers eux, encourager la revalorisation des métiers méprisés mais largement pourvoyeurs d'emplois. Il nous faut encourager une définition fine et prospective des besoins des territoires et une gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences. Je connais pour cela un outil formidable, madame la ministre, créé par Jean-Louis Borloo, nouveau compagnon de route de votre gouvernement : les maisons de l'emploi et de la formation, les MEF. Elles ne sont pas redondantes avec l'action de Pôle emploi ni avec celle des services de l'État, comme vous l'avez affirmé. Au contraire, elles en sont intrinsèquement complémentaires. quelques chiffres afin de démontrer, si besoin est, la pertinence de cet outil : 116 maisons de l'emploi portées par 10 354 communes pour 21 millions d'habitants concernés et plus de 1,5 million d'entreprises partenaires. l'emploi, au service de 4 400 communes, ont accompagné, l'an dernier, 100 000 personnes très éloignées de l'emploi dont 45 % ont trouvé un emploi durable- soit près d'une personne sur deux, madame la ministre 436 facilitateurs de la clause sociale d'insertion, pour la plupart formés par le réseau Alliance Villes Emploi- que je félicite ici pour son travail de fond -, ont développé plus de 11 millions d'heures d'insertion en 2016, soit 30 000 personnes recrutées- dont 72 % dans un emploi durable au bout de 24 mois.

Que représentent 21 millions d'euros sur un budget total de 15,3 milliards d'euros de crédits de paiement ? D'autant que vous pouvez mobiliser les maisons de l'emploi pour mener à bien votre plan d'investissement dans les compétences, le PIC. Vous pouvez également mobiliser les maisons de l'emploi dans le cadre de la politique de la ville.

Ledru-Rollin, devant la Constituante, défendait, dès 1848, le droit au travail : « On a dit, le droit au travail, c'est le socialisme. Je réponds : non, le droit au travail, c'est la République appliquée ». madame la ministre, appliquez la promesse de la République. Faites confiance aux acteurs locaux et aux entreprises. Donnez des gages aux élus des territoires en réinstaurant ce dialogue local et ces crédits aux maisons de l'emploi Si ces gages ne sont pas donnés, en l'état actuel de la mission, vous ne nous laisserez pas d'autre choix que de voter contre votre budget. La

voilà quelques semaines, l'INSEE confirmait les effets de la reprise économique en cours, avec 240 900 emplois salariés créés en un an, malgré un léger ralentissement au troisième trimestre de 2017.

structurelle majeure de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, avec pour objectif de réduire le taux de Les crédits de la mission « Travail et emploi » que nous examinons aujourd'hui sont indissociables de ces réformes, ainsi que des mesures générales de réduction du coût du travail inscrites dans Ce nouveau contexte justifie les orientations du budget de l'emploi pour 2018 dont les crédits seront de 15,2 milliards d'euros en crédits de paiement, et de 13,7 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Il recentrer l'intervention et le soutien de l'État sur les publics et territoires qui en ont le plus besoin. Ensuite, et surtout, il faut agir sur l'emploi durable en investissant dans les compétences, en priorité pour les personnes peu qualifiées. Le plan d'investissement dans les compétences sera ainsi doté de 15 milliards d'euros sur cinq ans. Dès 2018, 500 millions d'euros sont consacrés au démarrage de ce plan, en particulier pour la montée en charge de la garantie jeunes. Enfin, il faut accompagner les acteurs économiques dans l'anticipation et la gestion des transitions économiques. Le groupe La République en Marche partage entièrement ces priorités et orientations, ainsi que leur traduction dans les quatre programmes composant la mission dont il votera les crédits. Sans entrer dans le détail de chacun de ces programmes, quelques points méritent d'être soulignés. S'agissant du programme 102 « Accès et retour à l'emploi », le choix assumé par le Gouvernement sera de recentrer les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés spécifiques, tels les travailleurs handicapés. Ainsi, à la différence des contrats de génération, les emplois aidés seront maintenus à hauteur de 200 000 contrats dans le secteur non marchand en 2018, pour 1,46 milliard d'euros. Priorité sera donnée aux jeunes en insertion et aux chômeurs de longue durée, aux territoires ultra-marins et ruraux, ainsi qu'aux secteurs de l'urgence sanitaire et sociale et à l'accompagnement des enfants handicapés en milieu scolaire. Cet été, le choc a été d'autant plus difficile à surmonter que nombre de collectivités et d'associations, peut-être ingénument, n'avaient pas anticipé que seuls 280 000 contrats aidés avaient été budgétés en 2017, contre 459 000 en 2016. La diminution programmée des emplois aidés pour donner la priorité à la formation professionnelle est une stratégie que nous soutenons. convenons qu'une décrue plus progressive et laissant du temps à la pédagogie n'aurait rien gâché. S'agissant toujours du programme 102, nous tenons à souligner les efforts budgétaires réalisés pour la garantie jeunes, pour l'insertion par l'activité économique avec 5 000 nouveaux postes conventionnés,

Enfin, ce programme intègre la nouvelle action n° 03, Plan d'investissement des compétences, axée sur la garantie jeunes pour 2018, avant de monter en charge au fur et à mesure du déploiement du PIC. Il y a en effet urgence à insérer les 1,8 million de jeunes en situation de grande précarité qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation. Le coût total du dispositif pour 2018 est de 514,6 514,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 503,27 millions d'euros en crédits de paiement. S'agissant du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », je souhaite insister sur l'importance de l'action n° qui vise principalement à soutenir le développement de l'alternance, des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Ces crédits sont stables en 2018 et ceux du compte d'affectation spéciale progressent de 59 millions d'euros en 2018, dans l'attente de la réforme de l'apprentissage et de l'alternance, dont je ne saurais trop souligner l'importance fondamentale : il faut simplifier, dynamiser, disons-le, il faut rendre « sexy » cette voie d'accès à la vie active qui est aussi une voie d'excellence. J'attends donc avec impatience les crédits pour 2019 et pour les années suivantes. Madame la ministre, moi qui suis Européenne convaincue et élue du Haut-Rhin, je ne peux que conclure par un plaidoyer pour les échanges européens et la mobilité des apprentis. Le programme Erasmus est, à juste titre, un trentenaire acclamé. Son petit frère, « Erasmus plus », ne demande qu'à connaître la même destinée, pourvu que la volonté politique lui donne des ailes. Jean Arthuis car les législations du travail sur les apprentis diffèrent grandement au sein de l'Union. Notre jeunesse européenne mérite un tel effort, car elle a besoin du ciment qui la tiendra « unie dans la diversité », comme le proclame la devise de l'Union. La

Vous avez indiqué, madame la ministre, que ce budget marquait votre volonté de rénover profondément le modèle social. Il s'inscrit effectivement dans une logique globale de transformation du modèle social, dans le droit fil des contre-réformes du code du travail que nous avons combattues et de celles annoncées sur l'assurance chômage, sur les retraites et sur l'apprentissage. La baisse des crédits de la mission « Travail et emploi » est essentiellement due à la réduction de moitié du nombre de contrats aidés, pour une économie de 1,4 milliard d'euros environ.

Certes, la baisse du nombre de contrats aidés avait été engagée dans la loi de finances précédente, mais vous la poursuivez, alors que les effets négatifs commencent à se faire sentir sur le terrain. Le sentiment d'incompréhension des

il faut parler aussi de la colère légitime des maires, placés brutalement devant le fait accompli, cet été. Le Président de la République a reconnu lui-même, devant le congrès des maires, que les collectivités n'avaient pas été « dûment concertées ». Il avait ajouté vouloir maintenant qu'elles le soient Je vous pose la question, madame la ministre : où en est la concertation avec les collectivités et les représentants des associations ? Quelles solutions de fond et quelles alternatives proposez-vous si vous persistez dans votre intention de supprimer ou de diminuer fortement les contrats aidés ? Entendons-nous bien, je ne défends pas ici le ni la ni la généralisation de l'emploi précaire- ce ne serait pas dans les gènes des communistes. Des abus ont pu être commis, les résultats en termes d'insertion durable dans l'emploi

des contrats aidés du secteur marchand ont débouché sur un emploi au bout de six mois, ce taux atteint tout de même 41 % pour le secteur non marchand. Nous savons combien ces possibilités d'insertion étaient vécues

et non supprimé, surtout que vous ne proposez pas d'alternative pour ces centaines de milliers de bénéficiaires exclus sans ménagement de ce dispositif

... Alors que vous supprimez des moyens d'insertion existants, la concrétisation du plan d'investissement dans les compétences, pourtant largement médiatisé, se traduit à peine dans ce projet de loi de finances pour 2018 par rapport à l'enveloppe budgétaire. La réalité, c'est que dans un contexte de chômage de masse, au milieu de réformes plus globales visant à flexibiliser

c'est la politique de l'emploi dans les territoires qui est aussi mise à mal. De même, vous stabilisez les crédits de fonctionnement des missions locales, alors que vous prévoyez, plus de 15 000 entrées nouvelles dans le dispositif garantie jeunes. L'austérité dans les ministères touche aussi maintenant les opérateurs de l'État. Je pense au service public de Pôle emploi dont la subvention pour charges de service public diminue de 50 du redéploiement d'agents vers des services aux employeurs, ce qui pose la question de l'accueil et de l'accompagnement des privés d'emploi, notamment les plus en difficulté ? Comment ne

étonnant paradoxe tout de même, au coeur des priorités de notre pays, de constater cette diminution de crédits accompagnée d'une chute majeure des autorisations d'engagement, en recul de 2,7 milliards d'euros, à 13,7 milliards Paradoxe plus inquiétant encore quand la programmation triennale prévoit une réduction de budget à 12,89 milliards d'euros en 2019, puis à 12,57 milliards en 2020.

permettre à 100 000 jeunes d'y accéder. Ce dispositif, qui ouvre la voie à une intégration sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif et personnalisé, apprécié dans ses objectifs comme dans sa mise en oeuvre par les missions locales, est programmé à 514,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 503,27 millions d'euros en crédits de paiement,

entre une hausse de plus de 17 % des bénéficiaires et une baisse de 9 % des crédits ? Nous serons attentifs à votre réponse. notre pays, 780 entreprises adaptées apportent une réponse efficiente au chômage des personnes en situation de handicap, employant 27 000 d'entre elles, sur un total de 35 000 salariés. Elles bénéficient de deux aides : une aide au poste compensatoire du handicap du salarié et une subvention spécifique destinée au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée. de loi de finances pour 2018 prévoit d'augmenter le nombre d'aides au poste de 23 036 à 24 036 équivalents temps plein,

d'euros. Ces propositions non seulement méconnaissent la réalité de l'entreprise adaptée, mais vont fragiliser un certain nombre de structures et sont contraires aux engagements de l'État

Vive interrogation, encore, sur la création de 10 000 emplois francs dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par une aide différenciée suivant le type de contrat, avec une période expérimentale en 2018 et en 2019. Comment un dispositif non ciblé en termes d'âge ou de niveau de qualification pourrait-il ne pas entraîner un fort effet d'aubaine ? France Stratégie recommandait en 2015 « de restreindre le dispositif aux habitants les moins qualifiés pour éviter les effets de dépréciation des plus diplômés ».

à votre approche du dossier des contrats aidés, leur diminution ou suppression pour 2018 et la chute de 70 % à 50 % du taux de prise en charge par l'État. Je l'illustrerai en parlant du ressenti de la situation dans mon département, l'Aisne, parmi les plus foncés- hélas ! -sur les cartes du chômage, mais où la détermination des élus, acteurs associatifs ou économiques est totale pour rapprocher de l'emploi les habitants les plus en difficulté.

Ce sont des emplois socialement, économiquement, humainement indispensables quand, ici, leur disparition met en danger un organisme caritatif qui rayonne dans tout le département et distribue chaque année l'équivalent de plus de trois millions de repas elle met en danger des services de restauration ou de transport scolaires. L'annonce de l'été, c'est aussi un coup de massue, l'opprobre jeté sur des personnes souvent inscrites depuis plus de douze mois à Pôle emploi, allocataires de minimas sociaux, confrontées à divers handicaps de la vie pour lesquelles l'emploi aidé représentait un rôle dans la société, une dignité retrouvée, plus d'estime de soi. Cette dimension humaine est sans commune mesure avec les statistiques. D'autant plus quand la DARES, en novembre dernier, indique que 43 % des personnes sorties d'un contrat initiative emploi et 66 % des personnes sorties d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi sont en emploi six mois après la fin de l'aide.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le taux de chômage dans la zone euro a poursuivi sa baisse en octobre 2017 pour atteindre 8,8 %, mais il est encore de 9,5 % en France. Malgré la reprise de l'activité, nous sommes donc encore loin de la moyenne européenne. Derrière ces chiffres, ce sont des millions de Françaises et de Français qui souffrent au quotidien et qui réclament des solutions concrètes à ce mal français. crédits de cette mission doit donc être pour nous l'occasion de réviser, sans tabou, des dispositifs dont l'échec est avéré et dont le coût pour les finances publiques est trop élevé. Dans ce contexte, un effort important sera consenti sur les crédits de la mission « Travail et emploi » en 2018. Un effort, cela a été dit, de plus de 4 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 2 milliards d'euros en crédits de paiement. Malgré cette importante diminution, les crédits de la mission « Travail et emploi » seront maintenus à un niveau élevé. Je salue les efforts de pédagogie du rapporteur spécial, Emmanuel Capus, qui nous a démontré que les efforts consentis s'accompagnaient d'un redéploiement bienvenu de crédits vers les dispositifs qui fonctionnent. Je voudrais d'abord revenir sur la baisse de l'enveloppe consacrée aux contrats aidés 200 000 contrats dans le secteur non marchand seront conclus en 2018, entraînant une baisse de plus de 1 milliard d'euros par rapport à 2017. Ces emplois peuvent s'avérer utiles dans l'instant pour certaines collectivités territoriales et pour le secteur associatif. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'ils sont par nature des contrats précaires, subventionnés, et donc une réponse de court terme à la catastrophe nationale que constitue le chômage de masse. réponse qui, parce qu'elle est payée par le contribuable, sacrifie la croissance à long terme, et donc l'emploi. Nous déplorons ainsi que, pour les raisons politiciennes que nous connaissons, le précédent gouvernement ait tout fait pour droguer les collectivités aux contrats aidés. Dans ma mairie, j'ai toujours refusé de céder à cette ivresse encouragée par l'État, sachant pertinemment que le retour au réel n'en serait que plus douloureux pour les personnes concernées, les collectivités, les associations et le pays tout entier. Nous y sommes Malheureusement pour lui, madame la ministre, le gouvernement actuel paie, parce qu'il commence à les réparer, les erreurs du gouvernement précédent. Quoi qu'il en soit, le temps est venu de trouver des solutions durables pour l'emploi de nos concitoyens. de nos concitoyens. Par ailleurs, nous approuvons le choix du Gouvernement de se tenir à l'enveloppe votée par le Parlement. Jusqu'alors, l'enveloppe consacrée aux contrats aidés était systématiquement dépassée. Il faut saluer une décision courageuse qui participe de la sincérité globale de ce projet de loi de finances. J'en viens à l'autre point important de cette mission : la diminution de la subvention pour charges de service public versée à Pôle emploi. Celle-ci devrait passer de 1 507 millions d'euros en 2017 à 1 457 millions d'euros en 2018. comme l'a montré le rapporteur spécial, cette diminution devrait être compensée par une hausse plus que proportionnelle de la contribution de l'UNEDIC. Cette baisse ne devrait donc pas avoir d'impact significatif sur l'activité de Pôle emploi. Je passerai sur la suppression de dispositifs dont l'échec était patent, tels que le contrat de génération ou l'aide à l'embauche à destination des PME. Ils illustrent une fâcheuse habitude de nos politiques de l'emploi de privilégier des dispositifs coûteux et qui échouent à trouver leur public. Il nous semble, au contraire, que l'accent mis sur la formation dans ce projet de loi de finances est une bonne orientation. Ce plan se décline en deux volets principaux : tout d'abord, le renforcement de la garantie jeunes, avec un soutien accru aux missions locales pour assurer l'accompagnement de 100 000 jeunes la mise en place d'un plan de formation à destination des demandeurs d'emploi peu qualifiés et des jeunes en décrochage scolaire. Ces actions vont dans le bon sens et seront complétées avec profit, nous l'espérons, par les grandes réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui arriveront dans quelques semaines. Notre groupe et cette assemblée seront au rendez-vous d'un tournant nécessaire pour faire face aux mutations du monde du travail. Nous regarderons d'un oeil favorable une politique qui favorise la montée en compétence de l'ensemble des travailleurs tout au long de leur carrière, l'adaptation rapide aux transformations technologiques et la revalorisation de l'apprentissage. En attendant les débats sur ces questions fondamentales, le groupe Les Indépendants- République et Territoires votera ces crédits en l'état. Ils annoncent un redéploiement pertinent des efforts financiers de l'État vers les dispositifs les plus efficaces

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

la totalité en 2019. Ce projet de réduction des aides aux maisons de l'emploi est une catastrophe qui va amener ces structures à des fermetures définitives. Elles réalisent pourtant un travail qu'aucun autre acteur du service public de l'emploi n'effectue, comme l'a souligné M. Vanlerenberghe. Leurs missions ne sont pas redondantes, bien au contraire. Elles apportent un éclairage supplémentaire, tant d'un point de vue économique- accompagnement des entreprises sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, remontées des besoins locaux pour bâtir le programme régional de formation, création d'entreprises, clauses d'insertion -que d'un point de vue d'ensemblier territorial. Les maisons de l'emploi animent, coordonnent, supervisent, sont des acteurs centraux avec une bonne connaissance du terrain.

notre collègue Nathalie Delattre l'a très justement rappelé. Elles sont complémentaires de Pôle Emploi et lui apportent de réelles solutions. En particulier, leur raison d'être est dans l'initiative locale ; elles sont généralement bien pilotées, au même titre que les missions locales, par les élus locaux. Elles déclinent donc des actions qui collent au plus près des problématiques de notre territoire,

L'année dernière, j'avais plaidé, à cette même tribune, par souci d'une meilleure efficacité, pour une mutualisation des bases de données entre les opérateurs du champ de l'emploi. Les MEF et Pôle Emploi agissent en parallèle sur le même segment d'activité, mais sans avoir toujours développé de véritables synergies. L'échange de bases de données aurait été un levier d'amélioration : Pôle emploi possède une meilleure base de données, mais souffre, comparé aux MEF, d'une moindre efficacité opérationnelle. Il aurait été utile de se pencher sur cette question et d'améliorer les partenariats, au lieu de casser cet outil de proximité. Rappelons que les MEF réussissent à réunir autour de la même table préfets, élus, syndicats, chambres de métiers et Pôle Emploi, et peuvent ainsi proposer des solutions « sur mesure » au bassin d'emploi. Madame la ministre, que sont ces 10 millions d'euros au regard des presque 6 milliards d'euros de budget de Pôle emploi ? Cette mesure ne signe-t-elle pas la disparition programmée de la quasi-totalité des maisons de l'emploi, à laquelle il faudrait donc se préparer ?

pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, les associations familiales, bref, tout un tissu local d'intervenants qui utilisent ces contrats aidés afin de maintenir un niveau d'insertion économique et social en faveur de personnes souvent peu qualifiées et/ou éloignées du marché du travail. Les remettre en cause si brutalement, c'est prendre le risque de mettre fin à ces missions, ainsi qu'à des projets de cohésion sociale, sans les remplacer. L'effet est encore plus catastrophique en milieu rural. Cette annonce en cours d'année, au milieu du mois d'août, a mis le feu aux poudres. Mon collègue de l'Aisne, Yves Daudigny, a très bien décrit la situation dans notre département. Madame la ministre, vous n'aviez pas d'autre choix- c'est une bien mince consolation -que d'annoncer, en octobre, les domaines ciblés où ce qui reste de ces emplois serait désormais déployé, à savoir l'accompagnement des élèves en situation de handicap, l'urgence en matière sociale et de santé, notamment l'hébergement social et l'aide alimentaire, ceci en outre-mer et dans les communes rurales.

Pourquoi, madame la ministre, n'avez-vous pas décidé de reporter cette baisse drastique des contrats aidés à l'année prochaine, soit après les conclusions de cette mission, qui sont attendues pour la fin de cette année, au lieu de nous proposer un texte qui les supprime, ou presque ? Vous procédez à l'envers, et c'est bien dommage Concernant les orientations en faveur d'un véritable soutien à l'apprentissage, je veux, à titre personnel, souligner que les propositions du Gouvernement vont dans le bon sens. Je laisserai ma collègue Nicole Duranton développer ce point.

et les titulaires de ces contrats préféreraient travailler à temps complet, plutôt qu'à temps partiel- c'est bien évident. Mais ce que j'entends, sur le terrain, dans mon département du Pas-de-Calais, c'est : « Plutôt un contrat aidé que le chômage ! N'oublions pas que derrière ce terme de « contrat aidé », il y a des hommes, des femmes, des parcours, des vies. Retrouver du travail, c'est retrouver un cadre, des horaires, des échanges, une vie sociale et nous savons très bien que nombre de nos concitoyens ont ainsi pu renouer avec l'emploi et avec une vie digne. Ces mesures de réduction auront également un impact sur les communes, notamment sur les plus petites d'entre elles, qui pouvaient, grâce à ce dispositif, maintenir un service public de qualité alors même qu'elles sont victimes de la politique gouvernementale de réduction massive des dotations aux collectivités. Les associations, notamment celles qui mènent des actions de solidarité et d'utilité citoyenne, se trouveront elles aussi en difficulté pour assurer leurs missions. les élus que nous sommes pourraient vous démontrer qu'au-delà des clichés, les contrats aidés ne sont pas des solutions de facilité pour les communes et les associations qui profiteraient du système, mais bien des solutions humaines, qui sont proposées aux plus fragiles de nos concitoyens. Cette décision brutale et sans concertation démontre une méconnaissance totale du terrain et des publics concernés. En dépit de vos dénégations et de vos écrans de fumée, la finalité de cette mesure est bel et bien purement budgétaire, et les sénateurs socialistes et républicains ont déposé des amendements de rétablissement des crédits relatifs aux contrats aidés Concernant les crédits budgétaires pour l'insertion des travailleurs handicapés, depuis 2012, le nombre d'aides au poste financées par l'État a augmenté de 18 %.

Cette mesure permettra certes au Gouvernement de réaliser une belle économie, mais elle entraînera des difficultés financières pour nombre d'entreprises adaptées, qui devront licencier. Par ailleurs, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique va devoir réduire ses dépenses,

dites, mais nous pouvons tous, ici, nous accorder sur un constat : il est temps que notre pays remporte la bataille de l'emploi, qui nous préoccupe depuis près de trente Malgré nos sensibilités politiques différentes, nos appartenances partisanes diverses, nos territoires d'élection aux problématiques variées, ce combat est notre combat partagé, le combat de notre siècle. Une grande nation comme la France ne peut plus supporter que près de 10 % de sa population soit en situation de chômage ; une grande nation comme la nôtre ne peut plus accepter que près de 25 % des moins de 25 ans ne trouvent pas de travail ; une grande nation comme la France ne peut pas baisser les bras face à cette situation très grave. Depuis trop longtemps, nous reculons face aux réformes structurelles indispensables. Ce ne peut plus durer Dans notre société, accéder à l'emploi est synonyme de statut social. Je crois, à titre personnel, au rôle émancipateur du travail pour l'individu. Travailler, c'est sortir de chez soi ; c'est retrouver de la confiance, une estime de soi-même ; c'est, souvent, retrouver une dignité perdue à force de chômage et d'échecs. En France, nous avons pris la très fâcheuse habitude de toujours traiter le problème du chômage sous l'angle social : plus d'indemnités, toujours plus d'aides, comme si la puissance publique pouvait, à elle seule, combler le défaut d'embauche du secteur privé. Si le traitement social du chômage est une condition indispensable du respect de la dignité de nos compatriotes les plus fragiles, il ne doit plus constituer l'alpha et l'oméga de nos politiques en matière d'emploi. Madame la ministre, dans votre projet de budget, certaines mesures vont dans le bon sens. Je pense notamment au grand plan d'investissement en faveur de la formation que vous souhaitez mettre en place : oui, la formation des demandeurs d'emploi est aujourd'hui le point faible de notre pays. Toutes les études démontrent très bien qu'un chômeur formé, et de surcroît bien formé, a plus de chances d'accéder à l'emploi. En ce sens, la montée en puissance de la garantie jeunes, la formation des demandeurs d'emploi faiblement qualifiés ou encore la formation des jeunes « décrocheurs » constituent autant d'annonces intéressantes et ambitieuses, qu'il convient de saluer. la ministre, permettez-moi d'émettre des doutes quant à la réalisation de ces louables objectifs. Si l'on regarde de plus près la trajectoire budgétaire pluriannuelle que vous avez dessinée pour la période 2018-2022, on constate avec étonnement une diminution prévisionnelle des crédits alloués à la mission « Travail et emploi ». Je sais, madame la ministre, que l'État est un habitué de la formule « faire mieux avec moins » ; ce ne sont pas les représentants des collectivités territoriales que nous sommes qui vous diront le contraire. Mais je suis persuadée d'une chose. Si l'argent public ne règle pas tout, notamment en matière d'emploi, il a quand même une vertu sur laquelle nous pouvons nous accorder : il est la condition de la réalisation de politiques publiques ambitieuses comme celles que vous nous présentez. Je voudrais également revenir sur certaines annonces décevantes, qui soulèvent un certain nombre de questions. Je pense par exemple à la suppression de l'aide financière aux jeunes apprentis. Madame la ministre, l'apprentissage est une richesse ; il fait partie de l'ADN de notre pays. Depuis huit siècles, la France est le pays du compagnonnage, le pays de cette transmission technique et philosophique d'un savoir-faire artisanal et de valeurs symboliques fortes. La non-reconduction de l'aide financière à l'apprentissage constitue un signal profondément négatif à l'endroit de nos jeunes et des chefs d'entreprise de notre pays. Souffrant déjà d'un déficit d'image important, dû à des années de politiques discriminantes à l'égard des apprentis, et plus généralement des métiers dits « manuels », l'apprentissage, que vous comptez pourtant revaloriser, ne peut se développer sans dispositifs incitatifs forts. Pourtant, « l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit À l'heure actuelle, madame la ministre, aucune mesure nouvelle en faveur de l'apprentissage n'est contenue dans le projet de loi de finances. Le Gouvernement nous demande d'attendre un projet de loi annoncé pour le printemps 2018, sans que nous en connaissions encore les contours. les contours. Je peux, au nom de mon groupe tout entier, vous assurer de notre pleine vigilance sur ce sujet. En effet, nous croyons ardemment à l'apprentissage et à la nécessité de son développement partout sur le territoire national. Je regrette également, madame la ministre, la fin de l'aide à l'embauche à destination des PME, qui constituent pourtant le sel de notre économie, les forces vives qu'il convient de mobiliser si nous voulons gagner ensemble cette bataille pour l'emploi. J'ajoute à ce tableau le manque d'ambition de votre budget à destination de l'emploi des seniors, grand absent de ce projet de loi de finances pour 2018, alors même que les problèmes s'accumulent sans que nous puissions y répondre de manière claire et volontaire. Je voudrais enfin exprimer une inquiétude. Très attachée aux politiques d'inclusion, j'ai rendu en milieu d'année un rapport sur la culture et le handicap et préconisé, dans ce cadre, un certain nombre de mesures très concrètes pour faciliter l'accès des personnes handicapées à la culture. madame la ministre, que le rejet par l'Assemblée nationale de deux amendements qui visaient à sécuriser le financement de l'accès à l'emploi des personnes handicapées suscite chez moi une crainte réelle. Il est du devoir de l'État d'encourager massivement l'emploi des personnes en situation de handicap. Notre pays ne peut se satisfaire qu'un trop grand nombre de nos compatriotes, déjà profondément accablés par la maladie, se voient refuser un emploi au motif que les mécanismes d'incitation sont insuffisants. Veuillez conclure, ma chère collègue. Les personnes en situation de handicap doivent trouver toute leur place dans notre société. dans notre société. Pour conclure, madame la ministre, je veux vous faire partager une conviction profonde : votre gouvernement émet les bons diagnostics, notamment en matière d'emploi, mais ne se donne pas les moyens de remplir les objectifs qu'il s'assigne. Pour l'ensemble de ces raisons,

de vue, 2018 constitue un tournant important pour la mission « Travail et emploi », traduction budgétaire cohérente de notre volonté de rénovation profonde du modèle social français. de mieux protéger les salariés et de libérer les énergies des entreprises, afin que ces dernières investissent et créent de l'emploi, permettant au plus grand nombre d'accéder à l'emploi. La mission « Travail et emploi » reflète l'ambition des chantiers que nous avons engagés en ce sens.

Nous avons éteint une peur, et cette confiance nouvelle, liée à la reprise de la croissance, donne envie aux chefs d'entreprise d'embaucher ; les carnets de commandes se remplissent et la croissance repart avec robustesse-

stable de loi de finances en loi de finances, autour de 15,2 milliards d'euros, et en baisse assumée de 1,5 milliard d'euros à périmètre constant. Oui, il s'agit d'un budget de transformation ; il rompt clairement avec la logique de traitement statistique du chômage : nous basculons vers une politique d'insertion durable dans l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés, notamment les jeunes. Ce changement majeur se traduit par des choix assumés de réallocation de nos moyens. Premièrement, nous ferons un effort financier d'une ampleur sans précédent en faveur de la transformation des compétences incluant les formations qualifiantes et les compétences numériques, le plan d'investissement pour les compétences, qui sera doté de 15 milliards d'euros sur cinq de former et d'accompagner un million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et un million de jeunes décrocheurs à l'horizon de 2022. C'est un enjeu majeur : tous les experts, aujourd'hui,

%. Oui, le marqueur n° 1 du chômage, c'est le manque de qualification ! C'est pourquoi la compétence est la meilleure protection contre le chômage, et sera notre priorité. Ainsi, dans le cadre de ce plan d'investissement, dès 2018, nous engagerons un effort majeur dans la formation, avec 1,25 milliard d'euros en autorisations d'engagement et un triplement des crédits de paiement dédiés à cette politique.

Deuxièmement, nous mettons l'innovation sociale au service de la lutte contre l'exclusion sur le marché du travail. C'est le sens de la mission que j'ai confiée à Jean-Marc Borello, qui me rendra ses conclusions d'ici à la fin de l'année. Sa réflexion inclut les contrats aidés, mais son champ est beaucoup plus large. Dans ce contexte, les dispositifs d'insertion les plus efficaces seront soutenus et leur ciblage renforcé. Nous avons ainsi décidé d'accélérer nettement la création du dispositif dit des « emplois francs mettant en oeuvre cet engagement de campagne du Président de la République, qui permettra d'aider les personnes plutôt que les territoires, pour lutter efficacement contre les discriminations à l'embauche et l'assignation à résidence, dont sont victimes les diplômés comme les non-diplômés habitant dans les quartiers prioritaires de la

ans pour l'embauche en CDD d'un habitant d'un de ces quartiers prioritaires. C'est massif : c'est l'équivalent de neuf mois de salaire pour un emploi au SMIC. Nous avons ciblé cette mesure, à titre expérimental, pour 2018, sur cinq zones géographiques : la Seine-Saint-Denis tout entière, l'agglomération d'Angers, l'agglomération Val de France et celle de Cergy-Pontoise, dans le Val-d'Oise, le territoire Grand Paris Sud, qui englobe Grigny et Évry, et une partie importante des métropoles de Marseille et de Lille.

Par ailleurs, les 200 000 contrats aidés non marchands programmés pour 2018 pour un montant de 1,45 milliard d'euros seront réservés aux employeurs qui mèneront une véritable politique d'accompagnement et de formation, permettant de sortir durablement une partie importante de leurs bénéficiaires de la précarité.

en 2018 avec 822 millions d'euros. Si l'on compte également les exonérations spécifiques financées pour les associations intermédiaires et les chantiers d'insertion, l'effort de l'État sera supérieur à 1 milliard d'euros et permettra à 140 000 personnes environ d'être accompagnées dans leur parcours

Les dispositifs spécifiques aux travailleurs en situation de handicap s'établissent à ce stade à 377 millions d'euros, en hausse de 4 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour j'ai entendu les inquiétudes des représentants du secteur devant le projet de loi de finances, qui prévoit la création de 1 000 aides au poste avec une révision du mode de financement à compter du 1 juillet.

de leur engagement à une participation et de leur contribution à la réflexion sur les nécessaires évolutions des modalités de pilotage et de financement des entreprises adaptées. Aujourd'hui, le dispositif est très compliqué- il comporte notamment trois lignes budgétaires différentes -, ce qui ne permet pas aux entreprises adaptées, qui font un travail de long terme, d'avoir une visibilité suffisante. Nous devons réviser devons réviser ce mode de financement dans un sens plus efficace et plus durable. C'est le travail que nous avons engagé avec les entreprises adaptées. Nous devons aussi trouver les voies, par l'innovation notamment, du développement de l'emploi durable des personnes handicapées dans les entreprises adaptées comme dans les autres entreprises et voir comment les entreprises adaptées peuvent être un tremplin dans ce domaine. À ces conditions et au vu des travaux de concertation à conduire, je suis prête à reporter la mise en oeuvre de la réforme au 1 janvier 2019, alors qu'elle était initialement prévue pour le

se traduira par une augmentation de 8 millions d'euros des crédits dédiés au financement de ces aides au poste. Celles-ci seront ainsi financées selon les règles actuelles, dans l'attente des inflexions envisagées pour 2019. Ce besoin sera couvert en gestion sur les crédits du budget de l'emploi. les budgets de fonctionnement des missions locales, des EPIDE ou encore des écoles de la deuxième chance sont stabilisés à 285 millions d'euros. Le budget de l'AFPA est également stabilisé, à 110 millions d'euros. L'année 2018 L'année 2018 sera consacrée à définir une feuille de route stratégique à long terme de l'AFPA dont les bénéficiaires, les salariés et les partenaires de cette

La dotation de l'État à Pôle emploi évolue à la baisse, même si le budget total augmente de 20 millions d'euros, mais elle sera compensée par ses ressources dynamiques assises sur la masse salariale. L'année 2018 sera celle de la renégociation de la convention tripartite et pluriannuelle, et donc d'une vision de long terme du budget de Pôle emploi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avec la mission « Travail et emploi », notre triptyque « protéger, libérer, investir » est complet. Notre budget est sincère. Il nous permettra de saisir pleinement le potentiel du retour de la croissance

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », à hauteur de 750 millions d'euros, vers l'action n° 02, Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, du programme 102, « Accès et retour à l'emploi De manière brutale et sans concertation, le Gouvernement a décidé de ne financer que 200 000 contrats aidés en 2018, contre 310 000 en 2017 et 459 000 en 2016. Les contrats aidés sont d'une utilité sociale incontestable en permettant de répondre à des besoins sociaux dans les territoires : services à la personne et à la collectivité, éducation, santé, handicap. Ils permettent d'insérer et de former sur le long terme des personnes éloignées de l'emploi. En outre, leur coût est bien moindre que celui d'autres politiques publiques en termes de créations d'emplois. Alors que le coût annuel d'un emploi créé avec le CICE est estimé à 200 000 euros, que la prise en charge d'un contrat aidé par l'État pour un emploi d'avenir est estimée par la Cour des comptes à 11 000 euros par an et par jeune, celui d'un CUI-CAE s'élève en moyenne à 10 250 euros, toujours selon la Cour des comptes. Le présent amendement vise à intégrer un taux de prise en charge équivalent à celui de 2017.

Cette décision brutale s'est traduite par d'importantes difficultés pour les collectivités territoriales et les associations, pour lesquelles ces emplois étaient indispensables afin d'assurer dans de bonnes conditions certains services publics ou actions sociales. Une telle décision, prise sans concertation ni préavis, entraîne une véritable fragilisation de certains services publics, dans un contexte de diminution des dépenses : d'une part, certains emplois n'ont pas été reconduits ou ne le seront pas ; d'autre part, le montant qui sera pris en charge par l'État passera de 70 % à 50 %. De plus, ce choix jette l'opprobre sur les collectivités territoriales, soupçonnées de tirer profit de l'effet d'aubaine provoqué par ce dispositif pour bénéficier de financements complémentaires. Or la grande majorité des collectivités territoriales a atteint les objectifs fixés par le dispositif initial et mis en place une véritable insertion professionnelle des bénéficiaires de ces contrats. Cette décision a également mis à mal le tissu associatif, les associations concernées n'étant pas en mesure de recruter sans l'aide financière apportée par l'État. Les auteurs de cet amendement s'opposent à une telle décision dont les conséquences sociales seront dommageables, et ce malgré les domaines prioritaires identifiés par le Gouvernement sur lesquels seront ciblés les 200 000 contrats conclus en 2018, qui sont beaucoup trop restreints. En effet, outre leur utilité pour les collectivités territoriales et le tissu associatif de notre pays, ces contrats constituent des instruments importants pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. Les taux de sorties positives rappelés précédemment doivent ainsi s'analyser au regard du public concerné. Or, comme le souligne la DARES, « en 2015, 9 nouveaux bénéficiaires d'un CUI ou d'un emploi d'avenir sur 10 présentaient des difficultés particulières pour trouver un emploi C'est pourquoi cet amendement vise à augmenter de 214 102 016 euros le programme 102 de cette mission, plus précisément la sous-action n° 02.01, Insertion dans l'emploi aux moyens de contrats aidés.

Le secteur non marchand, en particulier le secteur associatif, subit une double baisse non concertée en 2018. Elle subit notamment une baisse du volume de contrats aidés, qui passent de 460 000 en 2016 à 320 000 en 2017, puis à 200 000 en 2018. Cette double baisse a de graves conséquences non seulement sur l'activité, mais aussi sur le modèle économique d'un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, parmi lesquelles les associations, intervenant auprès de publics fragiles ou encore sur l'employabilité et l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Le présent amendement vise à doter de moyens supplémentaires la sous-action Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés de l'action n° 02, Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Dans un contexte de rigueur budgétaire pour les collectivités territoriales et de chômage de masse pour les Français, les contrats aidés mettent en oeuvre un pacte gagnant-gagnant : ils permettent, d'une part, aux collectivités territoriales de pouvoir embaucher à coût avantageux, et donc de répondre efficacement à la mission de service public qui leur est confiée, et, d'autre part, aux personnes les plus éloignées de l'emploi de sortir de ce cercle vicieux qu'est le chômage. Enfin, le non-renouvellement d'une grande partie des contrats aidés aura un impact sur la mission de service public confiée aux collectivités territoriales. En effet, la suppression des emplois aidés amincira les marges de manoeuvre et l'autonomie financière des collectivités, au moment où nombre d'entre elles éprouvent déjà des difficultés à présenter un budget à l'équilibre. Celles-ci n'auront d'autre choix que d'effectuer des coupes budgétaires dans les différents services publics ou d'augmenter les impôts locaux. Par conséquent, les administrés verront, soit la qualité du service public s'affaiblir, soit leur feuille d'impôt s'alourdir. Le Gouvernement entend remettre en cause un outil primordial d'insertion dans l'emploi qui permettait de briser le cercle vicieux du chômage, sans concertation avec les acteurs sociaux concernés. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer un projet de loi de finances dont le mot d'ordre est l'injustice sociale et fiscale. Il prévoit ainsi de majorer de 40 000 la programmation des emplois aidants, à raison de 40 000 CAE supplémentaires pour 2018, ce qui permettrait

Premièrement, il s'agit d'une question de constance. En 2015, la commission des finances, suivie en cela par le Sénat, a souhaité la réduction du nombre de contrats aidés dans le secteur non marchand.

nombre d'arguments me paraissent peu adaptés au réel. Vous évoquez, en contrepartie de la diminution drastique des contrats aidés, l'élargissement du CICE la première année, puis la réduction des cotisations. cela ne concerne pas les mêmes structures ni les mêmes associations. Je ne doute pas que, dans les très grosses associations du secteur sanitaire et social, qui sont fortement employeur, la baisse de la masse salariale aura un impact positif.

La réduction de 40 % des emplois aidés en 2018 est inacceptable en ces termes. Certes, la mise en place de réflexions sur des évolutions relatives aux politiques de l'emploi, notamment pour nos concitoyens les plus éloignés du marché du travail et les moins diplômés, est nécessaire compte tenu des chiffres du chômage. Cependant, cette décision est contestable tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, il n'y a eu aucune concertation, ni avec le secteur associatif ni avec les élus locaux, ce qui est en contradiction totale avec l'accord de méthode convenu lors de la Conférence nationale des territoires, le 17 juillet dernier. Sur le fond, pour justifier ces suppressions, vous dénoncez le caractère coûteux et l'inefficacité de ces contrats en matière d'insertion professionnelle, et ce en ayant une lecture spécifique des données de la DARES. Beaucoup de ceux Beaucoup de ceux qui occupent un emploi aidé- emploi d'avenir ou contrat initiative emploi -ont de quoi être choqués par les propos tenus à leur sujet depuis des mois. Je souhaite m'adresser à eux aujourd'hui pour leur dire que leurs emplois sont utiles et qu'ils ont évidemment toute leur place dans notre société. Vous avancez un autre argument pour défendre la baisse du nombre de contrats aidés, que ma collègue Laurence Rossignol a évoqué, à savoir la transformation du CICE en baisse de cotisations dont bénéficieront les associations. d'abord, la diminution drastique du nombre de contrats aidés intervient dès cette année, alors que la transformation du CICE n'est prévue que pour 2019. Ensuite, la baisse des cotisations patronales ne sera pas équivalente à la prise en charge des contrats aidés, car nombre d'associations qui comptaient des emplois aidés n'ont pas de salariés. Il conviendrait aussi de cesser d'opposer contrats aidés et formation. On le sait, il n'existe pas de solutions miracles en matière de lutte contre le chômage, mais il y a une multitude de solutions pour faire face à des situations diverses. Pour les personnes les plus éloignées du marché du travail, chacun sait que le triptyque « accompagnement, formation professionnelle et entrée dans l'emploi » est indispensable. Au final, cette décision, qui s'apparente à un plan social massif, est une triple catastrophe : pour des milliers de salariés privés d'emploi, pour les collectivités territoriales empêchées d'assurer la continuité du service public de proximité, pour nos concitoyens privés des activités des associations, dont l'existence est aujourd'hui menacée.

qui irriguent le tissu local. Elles ont besoin de bénévoles, de femmes et d'hommes qui travaillent sur le vivre ensemble. Combien de petites associations, de petits concerts, de petites pièces de théâtre

l'ensemble de la collectivité, c'est-à-dire le monde de la cité et le bien commun tel qu'on le rêve aujourd'hui, peut être très

... Il en est ainsi décidé. La séance est suspendue.